Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi, tout d'abord, de citer le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat au sujet de l'article 8 : « Le présent article constitue une occasion sans précédent de modifier la structure de financement de la protection sociale au profit d'une part plus importante de la fiscalité et au détriment des cotisations sociales qui pèsent sur le travail et nuisent de ce fait à l'emploi et à la compétitivité des entreprises. »

mais prétendre que les cotisations sociales pèsent sur le travail et nuisent à l'emploi est proprement inexact. Les cotisations de sécurité sociale, parce qu'elles ont l'assiette la plus large possible, à savoir la production de l'appareil économique du pays sous toutes ses formes, ne sont aucunement nuisibles à notre compétitivité. Au contraire, elles y participent, parce que des salarié-e-s bien formé-e-s, bien payé-e-s et bien soigné-e-s constituent les meilleurs atouts d'une économie engagée dans la compétition mondiale. Les choix faits depuis des années et que vous confortez en les amplifiant- à savoir alléger les cotisations sociales d'employeurs de salariés travaillant, notamment, à temps partiel imposé

Et puis, vous qui traquez les économies sur les deniers publics, notamment à l'hôpital, cela ne vous pose-t-il pas de problème que, jusqu'en 2019, les entreprises bénéficient du versement du CICE dû au titre de 2018 et, en même temps, de réductions de cotisations pour la bagatelle de 24,8 milliards d'euros Et je ne parle pas des bénéficiaires du crédit d'impôt de la taxe sur les salaires, le CITS : leurs allégements de cotisations vont passer de 600 millions d'euros à 1,4 milliard d'euros chaque année, à compter de 2019 Pérenniser le CICE sous forme d'exonération de cotisations va à l'encontre de tous les travaux sérieux qui existent aujourd'hui sur ce dispositif et qui appellent plutôt à sa suppression. La parole

Nous le savons maintenant, le CICE n'est pas l'instrument le plus efficace qui soit : avec 100 000 postes créés ou préservés de 2013 à 2015, ses effets sur l'emploi ont été assez modérés. Les allégements de cotisations patronales qui interviendront en 2019 concerneront en priorité les bas salaires. C'est un moyen direct, supplémentaire, pour renforcer la compétitivité de la production française et favoriser l'embauche de nouveaux salariés.

Cette simplification profitera naturellement aux TPE-PME, qui consacrent trop de temps à se plier aux lourdeurs administratives. En leur facilitant ces tâches, nous les aiderons à créer des emplois productifs.

mais ce dispositif n'est pas durable, puisqu'il est imputé sur l'impôt, donc en décalage d'un an. Il est tout à fait cohérent de régulariser ce mécanisme une baisse des cotisations sociales, puisqu'il était assis sur la rémunération brute et que l'objectif premier était de baisser le coût du travail. Le Gouvernement a choisi

n'étant que transitoire, ne donne pas de visibilité aux chefs d'entreprise, tandis que la baisse des cotisations est durable. Pour l'année 2019, il faut noter que les entreprises bénéficieront d'un cumul du CICE et des exonérations de cotisations sera bénéfique pour les entreprises, mais creusera le déficit public. L'objectif est la création d'emplois, notamment pour les jeunes, dont le taux de chômage

L'article 8, tel que présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, vise à la transformation du CICE en un allégement définitif de charges sociales patronales. Le comité de suivi créé spécialement pour évaluer les effets du CICE vient de rendre son rapport pour la période allant de 2013 à 2015 : le bilan est assez éloigné des espoirs placés dans ce dispositif et surtout des grandes déclarations péremptoires du MEDEF

Le CICE devait servir à développer l'emploi, à favoriser l'investissement et à restaurer les marges des entreprises. S'il est vrai que les objectifs n'ont pas été totalement atteints, encore faut-il se laisser du temps pour pouvoir apprécier tous les effets

cause, vous nous proposez de transformer le CICE en un allégement de cotisations sociales, ce qui aura des conséquences potentiellement toxiques pour notre pays et notre protection sociale. Ainsi, rien ne garantit que la baisse du coût du travail sera utilisée pour investir, moderniser, innover ou renforcer nos armes

tout en renchérissant le coût du travail dans les secteurs employant des salariés qualifiés. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article et de jouer sur d'autres leviers pour stimuler notre économie.

En plus d'être coûteux, l'allégement de cotisations sociales ne garantira en rien que les entreprises bénéficiaires l'utiliseront pour créer ou préserver des emplois ou pour augmenter les salaires. Pis, cette mesure aura des conséquences sur le financement de la protection sociale et risque de devenir une trappe à bas salaires. Je m'étonne, madame la ministre, que le Gouvernement ne tire pas les leçons des erreurs passées et renforce, une fois de plus, ces aides non ciblées qui sont vouées à l'échec dans la lutte, pourtant essentielle, contre le chômage.

plus grande que la mienne ... J'ai simplement dit que le CICE n'avait pas atteint tous les objectifs qu'on lui avait assignés, qu'il fallait en tirer les enseignements et, par conséquent, faire en sorte que son octroi soit mieux ciblé et conditionné. Madame la ministre, je voudrais attirer votre attention sur les effets pervers

vise à faire la démonstration qu'une utilisation différente des recettes sociales est possible. Le manque à gagner engendré par le CICE et la suppression des cotisations sociales de la branche famille s'élève à 23 milliards d'euros, d'après le rapport de l'Assemblée nationale. L'échec du CICE et des exonérations sociales massives sans aucun effet sur l'emploi, ou presque, devrait nous conduire à

et de consacrer les 23 milliards d'euros ainsi économisés à la mise en place d'une véritable politique de protection sociale permettant notamment la suppression de la modulation des prestations

Aussi serait-il vivement souhaitable et juste de flécher cette baisse des charges vers les TPE et PME, qui sont souvent les grandes oubliées. En effet, si les grands groupes peuvent représenter des fleurons dans leur domaine, ce sont les très nombreuses TPE et PME françaises qui disposent des plus fortes capacités d'embauche. Il nous paraît donc nécessaire de réserver aux TPE et PME le bénéfice de l'allégement permanent de cotisations sociales, assorti, bien sûr, d'engagements en matière de création d'emplois.

en 2019, par un allégement de cotisations sociales patronales comprenant deux volets : un allégement de 6 points de cotisations sociales employeurs applicable pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC et un allégement majoré pouvant aller jusqu'à 9,9 points de cotisations sociales employeurs pour les salaires au niveau du SMIC,

En effet, toutes les études économiques ont démontré l'efficacité des politiques d'allégements de charges menées depuis les années quatre-vingt-dix lorsque ceux-ci sont concentrés sur les bas salaires. La réduction du coût du travail peu qualifié a un effet immédiat sur l'emploi. Il est nécessaire de concentrer l'effort sur les premiers niveaux de salaires, et non pas seulement sur le SMIC. Il faut savoir que, dans les entreprises, où les salaires et les charges peuvent représenter jusqu'à 80 % de la valeur ajoutée, la perte du CICE, couplée à la dégressivité de l'allégement de charges, aura inévitablement un coût. Or ce coût ne pourra pourra être répercuté totalement sur les contrats commerciaux, notamment auprès des clients publics, dont les budgets d'achat de prestations de services sont régulièrement revus à la baisse. incidence directe sur le coût du travail constitue une entrave à la compétitivité des entreprises et un frein à l'emploi, avec un risque de gel des embauches et d'incitation à geler également les salaires. C'est pourquoi il est ici proposé d'y remédier partiellement. Par ailleurs, le présent article Par ailleurs, le présent article fixe les modalités du dispositif d'allégement des cotisations patronales en remplacement du CICE. Or, pour les entreprises en décalage de paye, la suppression du CICE au 1 janvier 2019 signifie que le bénéfice du dispositif cessera fin novembre 2018.

et année sociale, il est proposé de synchroniser les deux dispositifs pour toutes les entreprises, y compris celles pratiquant le décalage de paye.

objectif qui semble tenir à coeur au Gouvernement. Nous proposons d'abroger l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, afin de supprimer les exonérations de cotisations patronales sur les bas salaires. Ces réductions dites « Fillon » ont été créées pour abaisser le coût du travail et inciter donc les employeurs à recruter à bas salaire, sans jamais augmenter par la suite la rémunération de leurs salariés.

coûtent chaque année 25 milliards d'euros aux caisses de la sécurité sociale. Il s'agit donc de la plus importante niche fiscale, pour reprendre les termes de la Cour des comptes. De façon plus générale, nous contestons la politique d'allégement de cotisations sociales à l'oeuvre depuis vingt ans. politique ruineuse pour les finances publiques, contribuant à tirer les salaires vers le bas. Quant à ses effets sur l'emploi, on ne peut que s'interroger sur leur réalité au regard du nombre de demandeurs d'emploi dans notre pays. La Cour des comptes relevait déjà, voilà dix ans, que « les nombreux dispositifs d'allégements de charges [étaient] insuffisamment évalués en dépit de la charge financière croissante qu'ils représentent[aient] pour les finances publiques ». Elle jugeait leur « efficacité trop incertaine pour ne pas amener à reconsidérer

aux limites prévues par l'arrêté du 20 décembre 2012, les employeurs sont autorisés à appliquer une déduction. C'est le cas pour les métiers du bâtiment ou les VRP, par exemple. La base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, qui inclut donc primes et avantages en nature, y compris les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels, qu'il s'agisse de remboursement au réel ou du versement d'une allocation forfaitaire. La déduction s'applique ensuite. Selon les annexes du PLFSS, l'abattement appliqué à la rémunération prise en compte au titre de l'allégement serait dorénavant réduit d'un tiers environ. Mathématiquement, le montant de la réduction, sur une assiette plus importante, serait donc moindre pour ces entreprises. Toutefois, il me semble que cette modification du calcul pour les entreprises pratiquant cette déduction forfaitaire spécifique est fondée sur un raisonnement erroné. En effet, à l'appui de cette disposition, l'annexe du PLFSS précise qu'un salarié rémunéré à hauteur

Par conséquent, non seulement les cotisations dues sont plus faibles, mais, en outre, l'exonération est applicable dans des conditions beaucoup plus favorables que celles du « droit commun ». Cet exemple ne tient pas compte de la réintégration des frais professionnels dans l'assiette de calcul. avant de pratiquer l'abattement, il faut ajouter au salaire les frais professionnels remboursés par l'employeur. L'assiette est donc, en réalité, forcément supérieure à 1,26

à rebours de la simplification souhaitée par le Gouvernement et chacun d'entre nous ici. En effet, elle va engendrer une complexification de la paie en créant une double assiette,

Monsieur Morisset, professionnels peuvent faire application d'une déduction forfaitaire de 10 %. Dans ce cadre, l'assiette de calcul des cotisations est constituée par le montant total des rémunérations et des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels, auquel est appliquée la déduction forfaitaire de 10 %. Par ailleurs, lorsque l'entreprise du bâtiment fait application de l'allégement général de cotisations sociales patronales, elle peut cumuler la déduction forfaitaire de 10 % avec celle-ci. Or, l'article 8 du projet de la sécurité sociale prévoit que le montant de l'allégement général de cotisations sociales patronales soit calculé sur une rémunération prenant en compte un taux de déduction forfaitaire spécifique réduit d'environ un tiers par rapport au taux de la déduction normalement applicable. conduirait à diminuer de plusieurs centaines d'euros par ouvrier du bâtiment le montant annuel de l'allégement général de cotisations patronales. Ainsi, pour un ouvrier rémunéré dans la limite de 1,6 fois le SMIC, entre l'actuelle formule de calcul et la nouvelle formule envisagée, la différence

remplacer le CICE. Or, pour les entreprises en décalage de paye, la suppression du CICE au 1 janvier 2019 signifie que le bénéfice du dispositif s'éteindra fin novembre 2018.

On le sait, les derniers chiffres disponibles font toujours état d'une différence très importante, en matière de salaires, entre les femmes et les hommes. Tous temps de travail confondus- temps partiels et temps complets -, les salaires des femmes représentent, en moyenne, 74,3 % de ceux des hommes. Autrement dit, les femmes touchent 25,7 % de moins que les hommes. Si une part de cet écart s'explique par le fait que les emplois à temps partiel sont très majoritairement occupés par les femmes, il n'en reste pas moins que, à temps de travail et à emploi occupé équivalents,

Cette discrimination sexiste a, de plus, un impact financier énorme pour le pays. Comme vient de le souligner la fondation Concorde, le manque à gagner pour l'économie française est évalué à 62 milliards d'euros par an

l'avouer, pas garantie. Un abattement d'assiette se traduit, certes, par moins de cotisations sociales, salariales comme patronales, mais aussi par moins de droits, notamment de droits à retraite. C'est d'ailleurs pourquoi la DFS ne peut en principe se pratiquer qu'avec l'accord du salarié.

Avec l'approfondissement des allégements généraux prévu par l'article 8, cet effet multiplicateur serait encore augmenté en 2019. L'article 8 ne neutralise pas totalement la DFS pour les allégements généraux, mais il permet, en renvoyant à un décret, d'éviter d'en accroître les effets multiplicateurs. Comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, dès lors qu'un effort très significatif

L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de charges spécifique pour les entreprises de services à la personne intervenant auprès des publics fragiles.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

peuvent être conduits à rejoindre un groupement associatif dont le siège social se trouve en dehors de la ZRR. L'objet de cet amendement est de maintenir, dans ce cas, les exonérations prévues

a pour finalité la justice sociale et pour objet une augmentation significative de la taxation des retraites chapeau les plus importantes. D'après la Fédération française des sociétés d'assurance, plus d'un million de Françaises et de Français sont concernés par ce dispositif. Dans la moitié des cas, les bénéficiaires perçoivent une rente inférieure à 2 000 euros par mois. Ce n'est évidemment pas ce public que notre amendement vise, mais bien certains dirigeants qui partent à la retraite en touchant des montants pharaoniques.

sont amenés à gérer des services d'aide et d'accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d'action sociale. Pour autant, ce rôle croissant n'est pas à ce jour pleinement reconnu, et les EPCI ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d'un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Cette différence de traitement est d'autant plus incompréhensible que les centres intercommunaux d'action sociale, les CIAS, bénéficient de cette exonération. Cet amendement vise donc à mettre fin à cette inégalité de traitement devant les charges sociales et à permettre de sécuriser le développement des coopérations intercommunales. Il s'agit non pas de créer une charge nouvelle, mais de constater que cette compétence est exercée également par les EPCI.

avait pour objet d'apporter des solutions aux difficultés de recrutement de vendangeurs. Les salariés employés sous contrat vendanges bénéficiaient d'une exonération de charges salariales, qui a été supprimée en 2014. Les charges salariales supportées par les vendangeurs n'encouragent pas les demandeurs d'emploi indemnisés à reprendre une activité temporaire, le gain de revenu pouvant être quasi nul. Ainsi, les difficultés de recrutement de vendangeurs sont toujours prégnantes. Cet amendement vise à rétablir l'exonération qui était en vigueur jusqu'en 2014. L'argument d'inconstitutionnalité invoqué lors de la suppression de l'exonération est contestable. En effet, dans un commentaire du Conseil constitutionnel sur la décision du 6 août 2014 portant sur la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 instituant une exonération généralisée des charges salariales sur les bas salaires, il est précisé une différence de traitement entre assurés d'un même régime placés dans la même situation peut être admise dès lors qu'elle repose sur des critères objectifs et rationnels et est en lien avec l'objectif poursuivi par le législateur le législateur ». L'exonération de cotisations salariales des travailleurs occasionnels viticoles vise à augmenter l'attractivité des contrats vendanges afin de faciliter le recrutement dans une période très resserrée. Les conditions de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et du salaire temporaire ne sont pas favorables au salarié, l'allocation d'aide au retour à l'emploi étant alors diminuée de 70 % du salaire brut. Adopter cet amendement permettrait d'encourager l'employabilité des personnes dans nos territoires et d'alléger les contraintes financières et administratives pour les viticulteurs. Une nouvelle fois, monsieur le ministre, l'occasion nous est donnée d'aider la ruralité

rectificative de la sécurité sociale pour 2014 visant à instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale a été censurée par le Conseil constitutionnel. Cela fait peser un doute sérieux sur le respect,

Aujourd'hui, plus que jamais, le secteur de la perte d'autonomie, qu'il s'agisse des aides à domicile ou des EHPAD, est à bout de souffle. Sur le principe, le groupe CRCE a toujours été opposé à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la CASA, car elle est supportée par les retraités, sont déjà fortement mis à contribution. Au travers de cet amendement, nous réclamons la création, en miroir de la CASA actuelle, d'une contribution de solidarité des actionnaires, au même taux de 0,3 %. Cette contribution permettrait d'abonder les comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Cette somme permettrait d'assurer une revalorisation des tarifs de l'aide à domicile

sommes, j'ose le dire, dans une situation d'urgence vitale : on ne peut pas laisser les personnes en perte d'autonomie, leurs familles, les salariés et les associations qui les emploient sans solution. L'aide à domicile est un secteur d'activité fondamentalement précaire, difficile, physiquement comme moralement, où les conditions d'exercice déterminent les conditions de vie des usagers et, parfois, leur vie tout court.

que l'avenant n° 35/2017 à la convention collective, qui prévoyait une augmentation très modeste de 0,44 % de la valeur du point au 1 octobre 2017, avait été refusé par la direction générale de la cohésion sociale.

à Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à supprimer la taxe sur les salaires dont sont redevables les hôpitaux publics en tant qu'employeurs. Cette taxe constitue une charge supplémentaire représentant entre 10 % et 12 % des dépenses de personnel, soit environ 4,25 % de l'ensemble des ressources hospitalières.

justifier que l'hôpital public soit mis à contribution, alors que les collectivités territoriales et les administrations publiques sont exonérées de la taxe sur les salaires

Évidemment, les hôpitaux ne se portent pas bien ; évidemment, nous devons transformer notre système de santé. Mais ce n'est pas en octroyant simplement des financements supplémentaires à l'hôpital public que nous remédierons en profondeur aux dysfonctionnements de notre système de santé.

L'assiette actuelle pénalise les entreprises d'achat-revente, qui supportent une fiscalité substantiellement plus lourde que les autres acteurs économiques, pour lesquels les achats consommés sont une composante mineure du chiffre d'affaires. C'est le cas notamment pour les agents commerciaux ou les commissionnaires, dont l'assiette est constituée de leur seule commission, ou l'ensemble des secteurs de la prestation de services. Cette inégalité de traitement n'est pas justifiée par la finalité d'origine de la C3S, qui est de compenser, par le biais de l'assurance maladie des indépendants, la perte de cotisations liée à l'application du régime général de sécurité sociale à une grande partie des dirigeants de société. Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les différents circuits économiques. Le système actuel altère de manière injustifiée la compétitivité des entreprises de négoce, qui assument tous les risques liés à la propriété des marchandises, tandis que les agents commerciaux ou les commissionnaires n'en supportent aucun. Par ailleurs, l'assujettissement à la C3S à chaque stade du circuit économique sans mécanisme de déduction aboutit à des doubles impositions et alourdit les charges des entreprises dans les circuits de distribution longs. Dans la perspective d'assurer une fiscalité équitable entre les modèles commerciaux traditionnels et les modèles commerciaux numérisés, il est indispensable de faire bénéficier les circuits traditionnels de conditions d'assujettissement à la C3S homogènes et de mettre fin à des disparités incitant les acteurs du circuit à

gratuites pour les grandes entreprises. Les PME, pour lesquelles ce taux est maintenu à zéro, ne sont pas concernées. La distribution d'actions gratuites au titre de la participation salariale avait été inscrite dans la loi Macron de 2015. Cette disposition avait pour objet de permettre à un créateur d'entreprise n'ayant pas les moyens de recruter un ingénieur, par exemple, d'attribuer à celui-ci des actions gratuites afin de l'intéresser au développement de la société. L'esprit initial a été dévoyé et ce dispositif a été étendu à toutes les entreprises du CAC 40, qui ne relèvent pourtant pas de la même logique. Aussi dans le projet de loi de finances rectificative de 2016 pour les grandes entreprises, tandis qu'un taux nul s'appliquait aux PME. Ce taux de 30 % n'a visiblement pas été dissuasif pour les entreprises du CAC 40, qui ont distribué 6,4 milliards d'euros d'actions gratuites au cours de l'année qui vient de s'écouler. La suppression de la quatrième tranche de la taxe sur les salaires représente déjà un cadeau de 120 millions d'euros pour les cadres des grandes entreprises gagnant plus de 150 000 euros par an. Le manque à gagner qui résulterait, pour les finances publiques, de l'abaissement du taux de cotisations patronales sur les actions gratuites distribuées par les grandes entreprises s'élèverait à 120 millions d'euros. Cela

la cotisation patronale de 30 % à 20 %. En 2016, les députés de la majorité ont voté un amendement visant à rétablir le taux de 30 %. Aujourd'hui, le Gouvernement souhaite ramener de nouveau à 20 % le taux des cotisations patronales sur la distribution d'actions gratuites pour les grandes entreprises.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

vise à étendre le régime d'exonération de la contribution définie à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale applicable aux routiers aux salariés des ports et des entreprises de manutention et à appliquer le forfait social de 20 %. tend à tirer la conséquence des accords sur la pénibilité des métiers portuaires. Aujourd'hui, le poids de la contribution spécifique menace la pérennité du régime et son application semble inappropriée au regard des spécificités de ces dispositifs. spécificités de ces dispositifs. Ce poids est d'autant plus lourd que les entreprises de manutention ont largement embauché pour compenser les départs anticipés. Il serait bon d'octroyer le même régime d'exonération défini pour les routiers aux salariés des ports et des entreprises de manutention, tout en les soumettant au forfait social unique.

l'avis de la commission ? La dérogation accordée au transport routier a vocation à être temporaire, le temps que les négociations pour la mise en place d'un système alternatif aboutissent. Il ne s'agit pas d'une dérogation qui pourrait être étendue à d'autres secteurs,

le dispositif d'exonérations de cotisations sociales pour les créateurs d'entreprise serait élargi à l'ensemble des créateurs et repreneurs d'entreprise dont le revenu annuel net est inférieur à 40 000 euros. Alors que ces exonérations sont actuellement réservées aux seuls chômeurs créateurs et repreneurs d'activité au titre de l'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise- ACCRE elles bénéficieraient désormais à tous les entrepreneurs qui commencent une activité. Cette réduction supplémentaire des cotisations sociales va encore déséquilibrer le financement de la sécurité sociale. Nous sommes d'autant plus dubitatifs que, selon une étude de l'INSEE de juin 2017, 30 % à 40 % des entreprises disparaissent au bout d'un an. La mesure prévue par le Gouvernement accélère ce mouvement et va donc dénaturer complètement l'ACCRE, pour avoir finalement un effet nul sur l'emploi. On voit bien la volonté de favoriser l'initiative individuelle, la course à la réussite, l'intention de devenir milliardaire, sur le modèle des entreprises américaines La réalité, c'est que l'immense majorité des individus qui deviennent leur propre employeur, en tant qu'indépendants, font une croix sur leurs horaires, leur salaire, leur vie sociale et leurs droits à la sécurité sociale. Est-ce que l'État doit favoriser cela ? Nous n'en sommes pas convaincus. Accompagner les créations d'entreprises au niveau régional en évaluant les besoins et les marchés potentiels et en accordant des facilités en fonction de critères environnementaux ou sociaux, oui ! Mais aider les indépendants à foncer dans le mur n'est pas notre vision de l'économie. Je rappelle encore les chiffres de l'INSEE de 2015, selon lesquels la moitié des autoentrepreneurs touchent moins de 500 euros par mois, soit bien moins que le revenu médian.

En début d'activité, les entreprises souffrent d'un manque de trésorerie. Ce dispositif permettra de consolider celle-ci, ce qui est très important pour l'avenir. Par ailleurs, cette réforme s'accompagne du doublement du chiffre d'affaires permettant de bénéficier du régime microfiscal.

Le présent article vise à mettre en place des mesures d'allègement de charges en faveur des travailleurs indépendants qui créent une entreprise en les exonérant de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de leur début d'activité. Compte tenu du fort taux de création d'entreprises outre-mer, et afin de pallier leur faible taux de survie, cet amendement vise à encourager la pérennisation de ces nouvelles activités dans le temps en augmentant la durée de l'exonération prévue par ce texte à deux ans, à titre expérimental, pour une durée de trois ans dans les départements d'outre-mer.

Actuellement, l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises, l'ACCRE, est cumulable avec le dispositif « jeunes agriculteurs ». Or la rédaction du présent article ne le permettrait plus dans l'avenir. Je tiens à rappeler que l'agriculture française traverse une crise durable et que, dans ce contexte, les questions du renouvellement des générations et de l'installation sont fondamentales. C'est pourquoi cet amendement tend à permettre aux jeunes agriculteurs bénéficiant de l'exonération

D'après les informations qui m'ont été transmises, ce cumul reste, à l'heure actuelle,

Monsieur Raison,

s'agit tout simplement de permettre à l'ensemble des jeunes qui veulent reprendre une exploitation ou s'installer de bénéficier des mêmes conditions et du cumul avec le schéma d'installation, tel qu'il existe aujourd'hui.

Celui dont je veux vous parler concerne la désertification médicale. En effet, c'est dans nos régions que l'on trouve la plus faible densité de médecins rapportés au nombre d'habitants. Ainsi en Martinique, 542 médecins seulement pour 100 000 habitants prennent en charge une population, qui plus est vieillissante.

ans. La répartition géographique des médecins demeure une inégalité difficile à enrayer. Les centres urbains connaissent une surpopulation médicale, alors que les campagnes pâtissent d'un manque criant de généralistes et de spécialistes. Cette mauvaise répartition géographique touche les zones qui souffrent

La mesure incitative expérimentale que nous proposons permettrait de rééquilibrer cette source d'inégalité qui touche souvent les zones les plus excentrées ou les plus difficiles d'accès et dans lesquelles la prise en charge médicale relève du service public à la personne. à l'esprit les propos du discours de Cayenne du Président de la République, qui affichait une ouverture totale à toute forme d'expérimentation prenant en compte les particularités du territoire.

Il est indispensable de proposer des mesures concrètes, avec un effet immédiat, car les constructions de pôles de santé et autres mesures, certainement intéressantes à moyen terme, ne suffiront pas à répondre à l'urgence que nous vivons dans nos territoires, notamment ruraux. Aussi, afin de conjurer cette situation, les auteurs de cet amendement proposent de créer une incitation pour que, à compter du 1 janvier 2018, les médecins retraités qui acceptent de reprendre ou de continuer un peu d'activité puissent cumuler leur activité libérale et leur retraite bénéficier d'une exonération de cotisations sociales jusqu'à 40 000 euros d'activité, ainsi que d'une exonération de cotisation foncière des entreprises. Ainsi, il serait clair pour les médecins qui s'engagent dans cette démarche qu'ils bénéficieront d'un revenu supplémentaire et à due proportion de leur activité. Par ailleurs, pour faciliter la mise en oeuvre de cette lutte contre la désertification médicale, nous proposons que les départements qui le souhaitent puissent organiser cette démarche sur leur territoire et se porter garants à l'endroit des médecins retraités volontaires de l'effectivité de ces mesures.

de la désertification médicale, mais c'est une affaire de justice sociale pour ces médecins. Au reste, nous avons intérêt à ce qu'ils puissent poursuivre leur activité dans l'espoir

qui concerne les médecins retraités,

compte tenu du trafic extrêmement difficile dans la conurbation centre, où se concentre l'essentiel de l'activité à La Martinique ? Je suis très déçue, parce que je suis sûre qu'une dizaine de médecins auxquels on attribuerait une

aux professionnels de santé qui exercent en secteur conventionnel et respectent les tarifs opposables. Je vous invite à ne pas fermer la porte à des mesures qui sont certes très sectorielles

d'entre nous. Madame Ghali, je regrette que vous laissiez entendre que je ne suis pas intéressée par ces enfants malades qui risqueraient de mourir dans les quartiers nord de Marseille. Votre argument ne tient pas : nous sommes tous convaincus ici

pour les entreprises de 5 salariés, pendant neuf ans. Ces mesures visent à maintenir l'emploi dans les territoires les plus fragiles, en créant des incitations à l'implantation des entreprises. Monsieur le ministre,

Or le principe d'une réforme du zonage des ZRR a déjà été décidé lors des deux comités interministériels aux ruralités qui se sont tenus en 2015, dans le prolongement d'une mission parlementaire. Ces nouveaux critères de classement sont justes et pertinents. Ils permettent de mieux tenir compte, dans une logique d'aménagement du territoire, de la fragilité des territoires ruraux. De plus, dans le cadre de la mise en oeuvre des allégements renforcés à compter du 1 janvier 2019- l'article 8 du PLFSS -, il est prévu de revoir l'ensemble des dispositifs d'exonération sociale zonés, dont les ZRR, qui deviendront moins favorables pour la plupart des salariés et dont, au moins sur le champ social, l'efficacité est fortement contestée par un rapport IGAS-IGF. Enfin, dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances pour 2018, un amendement a été adopté, permettant d'étendre jusqu'au 31 décembre 2019,

avec, comme point d'orgue, la signature de l'accord de Guyane du 21 avril 2017, qui engageait l'État sur le plan d'urgence et sur un certain nombre de mesures sectorielles. Parmi ces mesures, figurait la création d'une zone franche fiscale et sociale susceptible de favoriser l'attractivité du territoire et la croissance des entreprises qui y sont implantées. Si une mission d'expertise ministérielle s'est bien rendue en Guyane pour travailler sur ce sujet, les mesures transitoires prévues dans l'accord de Guyane n'ont pas été mises en oeuvre. Celui-ci prévoyait effectivement, pour 2017 et 2018, d'exonérer les entreprises guyanaises de cotisations patronales au titre de leurs salariés dont la rémunération est inférieure à 2,8 fois le montant du SMIC et de garantir ce niveau d'exonération pour les salaires dépassant ce seuil. Cet amendement vise donc à accorder cette exonération aux entreprises de Guyane pour l'année 2018, avant que la zone franche fiscale et sociale ne soit mise en oeuvre. Avec le déploiement du plan d'urgence, plusieurs chantiers d'infrastructure seront lancés au cours des trois prochaines années. Il est donc indispensable de permettre, dès 2018, le développement local par la relance de l'emploi et de l'investissement. Si toutefois l'exonération garantie jusqu'à 180 % du SMIC vous semblait trop importante, je vous proposerais, avec l'amendement n° 561, de garder les seuils existants, tels que prévus dans le code de la sécurité sociale, pour étendre uniquement la dégressivité jusqu'au

que le service était jusqu'à présent fermé à une liste d'activités et de services à domicile.